économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire Une disposition analogue figure à l'article L. 2241-9 issu de l'ordonnance n° 2017-1385, mais seulement au titre des dispositions supplétives. Nous proposons d'insérer la mention relative aux CDD et au travail temporaire dans la nouvelle rédaction de l'article L. 2241-1, parmi les dispositions d'ordre public. On constate en effet l'utilisation abusive et la répétition dans certains secteurs des contrats très courts, d'un jour ou deux. Une négociation au niveau des branches est nécessaire pour endiguer ce phénomène.

l'obligation de négocier au niveau de la branche passe, avec l'ordonnance, d'un rythme triennal à un rythme quadriennal. Pourquoi entériner ce recul, lorsque l'on connaît l'ampleur des inégalités salariales entre les femmes et les hommes hommes aujourd'hui ? Madame la ministre, dans un entretien accordé au vous avez fait connaître votre volonté de supprimer cet écart entre les femmes et les hommes d'ici à la fin du quinquennat. Pour y parvenir, il semble difficile de s'en tenir à un rendez-vous quadriennal

les entreprises françaises restent réticentes à mettre en place le télétravail, souvent en raison d'un cadre juridique jugé flou, notamment en matière d'accidents du travail, en dépit de l'adoption de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite « loi Warsmann Le recours au télétravail demeure faible en France par rapport aux pays scandinaves et anglo-saxons : le rapport rendu par les partenaires sociaux évoque une fourchette de 2 % à 6 % pour le télétravail le télétravail avec avenant et de 16 % à 20 % pour le télétravail informel. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, a complété les règles encadrant le télétravail en vue de le favoriser. Celui-ci devra désormais être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, d'une charte élaborée par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe. de cet amendement, le groupe du RDSE propose d'inclure le télétravail parmi les thèmes obligatoires à traiter lors des négociations collectives, en vue de susciter le dialogue social autour de cette organisation du travail qui intéresse de plus en plus les partenaires sociaux.

effet, négocier et faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes sans disposer des chiffres sur la réalité interne de l'entreprise ? C'est pourquoi, en nous fondant sur la pénalité prévue en cas de non-respect d'un accord sur l'égalité entre les femmes et les hommes, nous proposons de sanctionner à hauteur de 1 % de leur masse salariale les entreprises qui ne fournissent pas ces informations essentielles.

la commission a également émis un avis défavorable. En effet, son adoption ferait échec à la réforme visant à donner plus de liberté aux partenaires sociaux pour fixer la périodicité des négociations obligatoires de branche et aménager leur contenu, dans le respect de l'ordre public social.

La pénalité plafonnée à 1 % de la masse salariale vise actuellement deux cas de figure : l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes l'absence de plan d'action fixé unilatéralement par l'employeur. L'amendement vise à créer un troisième cas : l'absence d'informations sur la situation comparée des femmes et des hommes.

loi : la disposition adoptée oblige l'employeur à financer intégralement un expert pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle quand la base de données économiques et sociales ne comporte aucun indicateur sur ce thème.

opposable, ce qui constitue une grande nouveauté législative. Par ailleurs, les entreprises vont essayer de signer des accords et il y aura des chartes.

même si vous contestez cette analyse- j'y reviendrai -, l'ordonnance relative à la négociation collective prévoit de généraliser l'inversion de la hiérarchie des normes. La primauté de l'accord d'entreprise devient ainsi la règle, l'accord de branche

visait à instaurer des garde-fous sur la volonté de déroger, par accord collectif, à l'ordre public. Nous avons notamment à l'esprit le précédent de la signature par une fédération CFDT d'un accord fixant le salaire minimal dans la chimie en dessous du SMIC. Plus précisément, cet accord prévoit une augmentation des minima salariaux de 1,1 % pour l'année 2018, en deux temps, d'abord en janvier, puis en avril, alors que la revalorisation annuelle du SMIC, qui correspond à l'inflation, sera de 1,24

Bien sûr, on peut nous opposer des arguments, nous parler de garde-fous qui existeraient dans les textes, nous dire que, dans la mesure où l'on change les normes, il n'y a plus d'inversion de la hiérarchie des normes, par définition, puisque c'est la nouvelle loi qui s'applique.

demandons l'abrogation de ces dispositions et le rétablissement d'une véritable hiérarchie des normes, selon laquelle une norme d'un niveau inférieur ne peut déroger à une norme qui lui est supérieure.

mériterait sans doute d'être précisée. Je pense toutefois que la notion de « même cause » retenue dans l'amendement est source de complexité, tandis que celle de « même objet

En effet, vous refusez de reconnaître que le refus individuel d'un accord est susceptible de caractériser un licenciement économique et d'ouvrir les droits qui s'y rapportent. Selon vous, dans la mesure où le licenciement n'est pas contraint et rendu inévitable par les difficultés économiques de l'entreprise, comme dans le cas d'un licenciement économique, le salarié n'est pas tenu de bénéficier de l'accompagnement et de l'indemnisation prévus en cas de licenciement pour motif économique. En l'absence de cause économique, ces accords de compétitivité peuvent toutefois conduire à modifier les contrats de travail, donc à réviser les conditions d'engagement des salariés. Pour nous, une telle situation pose problème en tant que ce n'est pas au salarié qui refuse de voir ses conditions de travail modifiées par rapport à celles qui sont initialement prévues lors de son embauche de porter la responsabilité de son licenciement.

de notre rapporteur, marque l'élargissement des possibilités offertes à l'employeur d'utiliser l'emploi à tout moment et en toutes circonstances comme un instrument d'ajustement. Il ne s'agit pas d'une simple discussion sémantique. Nous relevons simplement que le mot « performance » s'applique à la seule entreprise concernée, tandis que le mot « compétitivité » implique l'existence de compétiteurs et la nécessité pour le salarié d'être à la hauteur pour maintenir l'existence de l'entreprise. Cette notion de « performance » exigée de chacun et de chacune d'entre nous, à tout propos et à tout moment, outre qu'elle démontre la pression exercée sur le monde du travail, ouvre pour l'avenir un champ élargi aux exigences des employeurs et aux menaces en matière de précarité et de licenciements. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression

de 1998, qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'informer et de consulter le personnel en cas de licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié. Or, en l'occurrence, le motif spécifique du licenciement

M. Jean-Louis Tourenne. Le code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de procéder au licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter les représentants du personnel. La directive 98-59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs oblige l'employeur à consulter les instances représentatives du personnel sur les mesures de reclassement prévues. La directive est claire : peu importe la nature économique ou non du licenciement ; dès lors que celui-ci est collectif, les procédures d'information et de consultation des salariés sont obligatoires. C'est pourquoi nous proposons de rétablir cette obligation dans le cas où dix salariés ou davantage refuseraient de se voir appliquer l'accord de compétitivité.

le Sénat a oeuvré en juillet dernier lors de l'examen de la loi d'habilitation pour que le licenciement d'un salarié qui refuse d'appliquer un accord de flexisécurité repose sur un motif qui ne soit ni personnel ni économique, mais spécifique et défini par la loi.

La commission a appelé « accord de performance sociale et économique » le nouvel accord de flexisécurité défini à l'article 3 de la première ordonnance. L'expression « accord de compétitivité », parfois utilisée pour le désigner, est en effet apparue impropre, non seulement parce que le nouvel accord peut avoir uniquement une visée défensive en cas de difficultés conjoncturelles ou structurelles, mais aussi parce qu'elle peut être source d'incompréhension chez certains de nos concitoyens. Je souhaite en outre rappeler à notre collègue Jean-Louis Tourenne n'a pas élargi le champ d'application de cet accord et que l'employeur ne peut pas unilatéralement l'imposer : il faut un accord avec les syndicats majoritaires. La commission émet donc un avis défavorable de l'amendement n° 150 me semble contradictoire : on ne peut pas, d'un côté, maintenir le motif spécifique du licenciement d'un salarié qui refuse d'appliquer l'accord de performance, et, de l'autre, appliquer les règles du licenciement économique quand plus de dix salariés sont licenciés.

Tourenne. Cet amendement vise à garantir le respect de la rémunération et du pouvoir d'achat des salariés. Il s'agit d'un amendement de précaution, dans la mesure où l'accord peut porter atteinte aux primes et accessoires de salaire en augmentant parallèlement le temps de travail et en le flexibilisant. : La parole est à M. Éric Gold. Cet amendement vise à rétablir le diagnostic partagé qui existait dans les accords offensifs, lorsque des baisses de salaires étaient envisagées. En effet l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a fusionné les accords de préservation et de développement de l'emploi et les accords de maintien de l'emploi en une seule catégorie, les accords dits « de compétitivité Ces anciens accords obligeaient l'employeur à transmettre les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic partagé, dès lors que la négociation portait sur l'aménagement de la rémunération. Or cette disposition ne figure plus au nombre des obligations de l'employeur dans le cadre des nouveaux accords de compétitivité. Si nous partageons cette idée que les accords de compétitivité doivent laisser toute sa place à la négociation collective, il nous semble toutefois opportun de rétablir le diagnostic partagé lorsque des baisses de salaires sont envisagées. Quel est l'avis de la commission

Ne réitérons pas les mêmes erreurs aujourd'hui ! J'ajoute que rien n'interdit aux négociateurs de maintenir la rémunération mensuelle des salariés lors de la négociation d'un accord de performance. La commission émet donc un avis défavorable l'amendement n° 170 rectifié, les accords de préservation et de développement de l'emploi, créés par la loi Travail, rendaient obligatoire le diagnostic partagé. Les syndicats pouvaient en outre recourir à un expert-comptable pour analyser le diagnostic de l'entreprise avec l'employeur avant d'établir un accord de maintien de l'emploi. Toutefois, nous avons tous pu constater depuis cinq ans que la multiplication des garde-fous juridiques était le meilleur moyen de tuer dans l'oeuf les accords de flexisécurité.

autour des modalités de préparation de cet accord apparaissent trop faibles. Ainsi, la nullité de l'accord qu'entraînerait l'absence de préambule a disparu. le préambule présente de manière succincte les objectifs visés. Il s'agit d'une sorte de note de synthèse, lisible par tous, qui permet d'améliorer la visibilité et la bonne compréhension des accords. L'intérêt pour les salariés et l'entreprise est évident : ils bénéficient ainsi d'une meilleure connaissance de la norme conventionnelle applicable. Si la loi de 2016 a prévu de ne pas sanctionner l'absence de préambule par la nullité des accords et conventions conclus, sauf si l'accord en décidait autrement, c'est pour éviter de faire peser une nouvelle obligation sur les organisations syndicales.

Il est indispensable de doter les partenaires sociaux de tous les outils permettant ce diagnostic partagé et d'améliorer la visibilité de tous les salariés.

pour les nouveaux accords de performance. J'ajoute que la sanction de la nullité me paraît quelque peu disproportionnée et que les négociateurs ont l'obligation de prévoir un tel préambule pour exposer les objectifs de l'accord de performance. Restons-en là ! La commission émet donc un avis défavorable l'avis du Gouvernement, Mme la ministre

On pourrait partager ce point de vue, sauf que la négociation telle que vous l'avez définie n'a pas les vertus que vous lui prêtez. Nous l'avons dit et redit : il n'y a pas de délégués syndicaux

dans la mesure où il existe une relation de subordination entre l'employeur et ses salariés. Dès lors, tout l'édifice que vous construisez risque de s'écrouler, madame

qu'il a été modifié à l'Assemblée nationale par le présent projet de loi, offre, selon la commission, des garanties suffisantes aux salariés qui refusent l'accord. Le principe étant désormais l'application automatique de l'accord collectif dans l'entreprise, y compris sur les stipulations contraires et incompatibles des contrats de travail, il n'est pas nécessaire de prévoir en plus des règles pour obtenir l'accord des salariés en cas de modification de leur contrat de travail. C'est incroyable ! La commission émet donc un avis défavorable.

à M. Jean-Louis Tourenne. Il existait quatre régimes différents, qui obéissaient à quatre procédures différentes, qui conduisaient à quatre motifs de licenciement différents et qui donnaient lieu à quatre modalités d'accompagnement différentes des salariés. L'article proposé par les ordonnances tend à harmoniser et à simplifier ces régimes, ce qui est tout à fait louable. Seulement, si le salarié refuse l'accord, on considère qu'il commet une faute et il peut donc être sanctionné par un licenciement. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour refuser l'accord. Ce délai, nouveau, nous semble trop court.

Je ne suis pas certain de saisir l'intention des auteurs de l'amendement. Aux yeux de la commission, et aux miens, le délai de réflexion d'un mois protège à la fois l'employeur et le salarié. Un mois de réflexion n'est pas excessif compte tenu des enjeux d'un tel accord et de ses conséquences en cas de refus du salarié. La commission demande donc le retrait de cet amendement

directe et automatique dans l'entreprise de l'accord de performance. Il n'est donc pas souhaitable de créer des règles spécifiques pour l'acceptation de l'accord. Ce sont les règles de refus qui doivent être définies, non pas celles d'acceptation. La commission émet donc un avis défavorable.

Tourenne. La possibilité de conclure de tels accords doit s'accompagner d'un droit à l'expertise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ce droit était inscrit dans les accords de préservation et de développement de l'emploi et financé par l'employeur. En fait, le problème, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, est que les ordonnances introduisent des dispositions qui visent- l'intention

Pourtant, la qualité du diagnostic analysé et partagé sur la situation de l'entreprise est indispensable en l'espèce et faciliterait sans doute les opérations éventuellement de compression du personnel. Sinon, comment les organisations syndicales et les élus du personnel pourront-ils disposer des informations indispensables pour déterminer leur position au regard des accords proposés ? C'est pourquoi nous proposons de réintroduire ce droit explicitement.

La création du conseil d'entreprise, qui donne des compétences de négociation aux élus du personnel, permettrait de répondre aux attentes des auteurs de l'amendement. La commission émet donc un avis défavorable

la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi ; les expertises sur les projets de licenciements collectifs pour motif économique ; en cas de risques graves constatés dans l'établissement. En revanche, l'employeur finance à 80 % et le CSE à hauteur de 20 %- sur son budget de fonctionnement -les frais d'expertise liés à la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise- depuis 2013

Cet article prévoit que les nouveaux accords sont « présumés négociés et conclus conformément à la loi ». En conséquence, il appartient à celui qui conteste leur validité d'apporter la preuve qu'ils n'ont pas été négociés ou conclus conformément à la loi. C'est une règle de base du droit. la mention portée dans l'ordonnance mérite deux observations. D'une part, nous sommes là dans le droit du travail, si tant est que vous le souhaitiez, pour le faire dériver vers le droit civil des obligations et le droit commercial de la prestation de service. Si donc le droit du travail a encore une autonomie, pourquoi la présomption de conformité à la loi d'un simple accord entre parties privées doit-elle être explicitement mentionnée ? S'agit-il de faire pression en cas de contentieux ou de dissuader de former un recours ? part, cette présomption ne nous paraît pas être une bonne chose dès lors que la base de données nationale rendant publics les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement prévue par la loi de 2016 n'existe pas.

Nous estimons que le délai de deux mois prévu pour le recours contre les accords collectifs est trop court, particulièrement en raison des nouvelles modalités de conclusion. Nous proposons donc de le porter à six mois. L'amendement n° Comme cela vient d'être dit, cet article valide tout accord ratifié au nom d'une présomption de légalité d'un accord d'entreprise majoritaire. Mais quand on sait que les négociations d'accords d'entreprise sont largement favorables au patronat, une telle mesure signifie que ce dernier pourra imposer sa « loi » en toute légalité, même si les mesures qui sont prises se révèlent illégales. D'ailleurs, dans un document publié le 7 juin dernier par le journal, la Direction générale du travail annonce clairement que cette présomption de légalité vise en fait à restreindre le contrôle du juge sur les accords collectifs. C'est clair ! L'ordonnance vise donc bien à éloigner les salariés des moyens de faire respecter leurs droits. Ainsi, les syndicats auront moins de temps pour analyser le contenu des accords et apporter la preuve d'une non-conformité de ces derniers avec la loi. Et même s'ils arrivent à le faire, ils ne pourront pas véritablement obtenir gain de cause, car le recours aux prud'hommes sera toujours à l'avantage de l'employeur, en raison, notamment, du plafonnement préalable des indemnités. La présomption de légalité, c'est donc donner un chèque en blanc pour que les employeurs enfreignent la loi et les droits des salariés. C'est tout simplement leur donner les pleins pouvoirs. C'est pourquoi nous demandons l'abrogation

En effet, cette disposition permet la modulation de l'annulation d'un accord collectif jugé illégal. Si un accord prévoyant une diminution de salaire est jugé illégal, l'employeur pourrait échapper

Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. En conséquence, il revient à celui qui les conteste de démontrer que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La chambre sociale a étendu cette jurisprudence aux différences de traitement entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle, puis aux différences de traitement résultant d'accords d'établissement au sein d'une même entreprise. La commission émet donc un avis défavorable

J'ajoute que les salariés conservent la faculté, qui n'est pas limitée dans le temps, d'attaquer indirectement, par voie d'exception, un accord devant le juge judiciaire quand il est lié à un litige individuel. La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement. la commission souhaite conserver les trois articles mentionnés dans cet amendement de suppression. Le premier article porte sur la charge de la preuve en matière de recours contre accord. Nous venons de le voir avec l'amendement n° 91. Le deuxième concerne le délai de prescription des actions en nullité, fixé à deux mois. Nous venons d'en parler avec l'amendement n° 92. Le troisième autorise autorise le juge à moduler dans le temps les effets de sa décision en cas d'annulation d'un accord, en reprenant une jurisprudence du Conseil d'État du 11 mai 2004,. Tous ces articles

n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit une obligation de formation, imposant à l'employeur des efforts de formation ou d'adaptation du salarié avant qu'un licenciement économique ne puisse intervenir. C'est très bien, mais cette obligation n'est aujourd'hui ni limitée ni précise. Il peut cependant être compliqué de former un salarié pour un poste disponible s'il ne dispose pas de suffisamment de compétences

la commission ? Cet amendement de notre collègue Daniel Chasseing vise à préciser que l'employeur n'est pas obligé de proposer des actions de formation de base aux salariés avant un licenciement économique. Il est vrai que la formation professionnelle doit, hélas, souvent pallier les carences de la formation initiale, mais cet amendement risque d'envoyer un mauvais signal, alors même que le Gouvernement veut mettre l'accent sur la formation tout au long de la vie. En outre, la notion de « connaissances de base » me paraît floue et

Alors que l'article 3 prévoit la fusion des instances représentatives du personnel au sein du nouveau conseil social et économique, le CSE, entraînant au passage la disparition des CHSCT, des comités d'entreprise et des délégués du personnel, cette fameuse ordonnance balai prévoit d'élargir la capacité de négociation du futur conseil d'entreprise. En effet, l'article 3 autorise les entreprises à transformer, par accord majoritaire avec les syndicats, le nouveau CSE en conseil d'entreprise, lequel pourrait même négocier des accords avec les employeurs. Par exemple, un plan de sauvegarde de l'emploi pourra être négocié par le conseil d'entreprise, et non plus par les organisations syndicales représentatives. En attendant de discuter de cette sixième ordonnance, celle dont nous débattons à cet article prévoit la disparition des CHSCT et leur remplacement par une commission « santé, sécurité et conditions de travail », mais uniquement

pour devenir des acteurs incontournables dans la prévention des risques professionnels, qu'ils soient physiques, chimiques ou organisationnels. Cette montée en puissance s'est faite, alors que se développaient des maladies psychosociales et et que les pathologies plus classiques se maintenaient à un niveau élevé. Malgré leurs limites, les CHSCT remplissaient une fonction spécifique, préventive, que vous prenez la responsabilité de supprimer. Pour notre part, nous nous opposons à cette régression, qui ne tardera pas- nous en sommes convaincus -à montrer des effets négatifs, et cela bien au-delà de l'entreprise.

des délégués du personnel, du CHSCT et du comité d'entreprise aura pour effet de relativiser les questions de santé au travail. Je l'avais dit l'été dernier ici même et je le redis aujourd'hui encore une fois, il s'agit d'une grave régression, notamment en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. On nous avait promis qu'une commission traiterait les questions d'hygiène et de santé et celles liées aux conditions de travail bénéficierait de la personnalité morale pour pouvoir ester en justice. Comme l'a fait remarquer Jean-Louis Tourenne, seules les entreprises de plus de 300 salariés seront obligées d'instaurer cette commission qui, d'ailleurs, n'aura pas de personnalité morale Et des autres entreprises ? Je veux encore rappeler que chacune des trois instances que vous voulez fusionner a une histoire, et surtout une raison d'exister. Elles permettent aux salariés d'intervenir et de s'exprimer. Par exemple, les CHSCT ont un rôle irremplaçable pour vérifier que les lois et règlements ayant un rapport avec la sécurité travail sont bien respectés. Ces comités sont aussi des lanceurs d'alerte dans le domaine de l'environnement et pour bien d'autres questions encore. Comme l'écrivait un sociologue du travail, les élus du CHSCT constituent la mauvaise conscience de l'employeur, lui rappelant sans cesse les conséquences de ses décisions sur les salariés. Voilà qui explique que certaines organisations patronales considèrent bon nombre de ses prérogatives comme exorbitantes. Le contre-pouvoir que constituent les CHSCT semblait en effet les gêner. « Cachons ces conditions de travail que nous ne saurions voir ! », pourrait-on dire pour expliquer cette position ... Je persiste fusionner toutes ces instances en une seule, c'est enlever de l'efficacité et de la force à chacune d'elles, à commencer par le CHSCT, dont le remplacement par une hypothétique commission dans les entreprises de moins de 300 salariés ne saurait suffire.

vote des lois dont le XX siècle n'a pas voulu. Et si le XXsiècle n'en a pas voulu, c'est que ces lois n'étaient pas fidèles aux promesses de justice de la République.

Qu'il s'agisse des revendications du quotidien, de la santé ou des conditions de travail, chaque élu a un rôle spécifique, tout en restant ancré dans la réalité de son entreprise. La création par ces ordonnances du comité social et économique détricote ce maillage au plus près de la réalité du travail et des salariés.

notre groupe ont dénoncé. Ensuite, la suppression du CHSCT en tant qu'institution autonome est très grave, car elle contribue à diluer les questions de santé au travail, qui sont pourtant fondamentales à l'heure où les techniques managériales augmentent les risques psychosociaux.

La suppression du CHSCT et son remplacement par une hypothétique commission dans les entreprises de moins de 300 salariés constituent, à notre sens, une régression grave

qui concerne la liberté du conseil social et économique de décider du transfert de l'excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles, le projet de loi de ratification revient sur un droit du CSE : selon les informations disponibles, ce transfert serait limité à 10 %.

des entreprises de moins de 50 salariés par l'association de gestion du Fonds paritaire national. Il est indispensable de prévoir la prise en charge de ces salaires sur la base d'un forfait, puisque l'association ne sera pas en mesure de connaître précisément la rémunération des salariés ayant participé aux

une atteinte à la protection des données personnelles. En outre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité de financement de missions d'information et d'animation de la formation économique, sociale et syndicale par la contribution des entreprises. En effet, à la suite à la concertation avec les organisations syndicales, il est apparu que la seule subvention de l'État ne pourrait couvrir durablement les dépenses relatives aux missions d'animation et d'information qui incombent aux organisations syndicales.

la prise en charge par le Fonds paritaire de financement du dialogue social de la rémunération des salariés des PME amenés à participer à des négociations au niveau de la branche. amendement vise à préciser qu'il s'agira d'une prise en charge forfaitaire, faute de pouvoir transmettre au Fonds des informations sur la rémunération de chaque négociateur. s'agit donc d'un ajustement technique et il appartiendra au Gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant de fixer ce forfait par arrêté. Par ailleurs, été complété, il y a quelques instants, pour réintroduire la possibilité pour le fonds paritaire de prendre en charge, au titre de la contribution des entreprises, la formation économique, sociale et syndicale. Cette modification ne modifie pas l'avis de la commission, qui reste favorable.

Le présent amendement a pour objet de permettre la mise en place du comité social et économique de manière anticipée lorsque les mandats des anciennes IRP arrivent à échéance entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019, qui n'est pas prévue par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Cet amendement vise également à prévoir que l'accord collectif et la décision de l'employeur permettant de faire coïncider l'échéance des mandats pour une mise en place du comité social et économique simultanée au niveau de chaque établissement puissent fixer des durées de mandat différentes pour chaque établissement distinct pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique.

Dans le cadre d'un accord, les partenaires sociaux de l'entreprise pourront s'entendre pour réduire la durée des mandats des élus actuels lorsque ceux-ci s'achèvent dans le courant de l'année 2019. De plus, ils pourront adapter la temporalité des comités d'établissement pour tenir compte des contraintes propres à l'entreprise. La commission

des contraintes dans l'entreprise et, ainsi, prétendument favoriser la compétitivité et l'emploi. Le présent amendement vise non pas à faire le procès des seuils sociaux, mais, à partir des éléments de constat et d'analyse qui seraient fournis par le Gouvernement, à ouvrir la voie à une harmonisation, voire à un lissage des différentes strates d'obligations, notamment pour améliorer l'efficacité du dialogue social, dans le droit fil de la création du comité social et économique. Les effets de seuil peuvent provoquer des comportements d'évitement qu'il convient de mesurer pour mieux les corriger. Quel est l'avis de la commission ? Il s'agit

puisqu'il comporte également une problématique fiscale ou encore de réglementation environnementale. En matière de représentation du personnel, la présente réforme apporte déjà des réponses aux difficultés rencontrées par les entreprises avec une instance unique à partir de 11 salariés, le franchissement du seuil de 50 salariés n'étant plus synonyme de création de deux instances supplémentaires. De plus, des aménagements sont apportés aux modalités de prise en compte du passage de ces seuils et d'application des obligations qui leur sont afférentes.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de préciser que, dans les cas où aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a recueilli 10 % des suffrages exprimés, qu'il ne qu'il ne reste plus aucun candidat ayant rempli cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit d'être désigné, le délégué syndical le délégué syndical peut être désigné parmi les anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au second alinéa de l'article L.

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à clarifier l'impact de la limitation à trois du nombre maximal de mandats de représentant du personnel pouvant être effectués par un élu sur la désignation des délégués syndicaux, qui doivent en principe avoir recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles. Il est prévu que, si aucun candidat n'a atteint ce seuil ou qu'il n'en reste plus dans l'entreprise, l'organisation syndicale pourra désigner un ancien élu ayant déjà effectué trois mandats. Il ne s'agit pas de contourner cette nouvelle règle, auquel cas je serais tout à fait opposé à cet amendement, mais de permettre aux organisations syndicales de s'y adapter et de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale, protégée notamment par la convention n° 87 de l'OIT. La commission a donc émis un avis favorable

en cas d'atteintes au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées à l'objectif.

très forte du droit d'alerte, l'intervention des délégués du personnel peut avoir, dans certaines circonstances, plus de poids qu'une autre. Alors que, jour après jour, l'actualité nous rappelle que des faits de harcèlement moral ou sexuel terribles se produisent dans tous les milieux, vous n'ouvrez le droit d'alerte au CSE en cas de danger grave et imminent que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Dès lors, une question se pose considérez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer au CSE un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes dans les entreprises de moins de 50 salariés ? Il nous paraît important de lever cette ambiguïté le CSE doit avoir le même droit d'alerte dans toutes les entreprises, qu'elles emploient plus ou moins de 50 salariés. Le présent amendement vise donc à rétablir ce droit d'alerte en cas d'atteinte aux personnes pour les représentants au comité social et économique dans les entreprises d'au moins 11 salariés. ? Les auteurs de cet amendement craignent que la création du CSE ne se traduise par la disparition du droit d'alerte des élus en matière d'atteinte aux droits des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés. Je tiens à les rassurer, leurs craintes sont infondées et leur amendement est satisfait, puisque, à la suite de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, puis par notre commission des affaires sociales, il est désormais bien précisé que la délégation du personnel du CSE dans ces entreprises exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59

Taillé-Polian. Nous pourrions croire à la bonne foi du Gouvernement sur son souhait de conforter la santé au travail dans les entreprises si ces commissions au sein des CSE avaient exactement les mêmes prérogatives que les CHSCT auparavant. Bien sûr, dans certaines entreprises de plus petite taille, ces commissions n'existeront plus ou ne seront pas obligatoires, mais, même là où elles existeront, il y aura des différences dans les prérogatives dont elles vont bénéficier, notamment en matière de prévention des risques et de vigilance sur le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité. L'objet de cet amendement est donc de réintégrer toutes les dispositions dont se prévalaient les CHSCT et de rétablir l'entière responsabilité de l'employeur en matière de prévention des risques, car nous pensons que cela permettra une meilleure implication de celui-ci

commission ? Selon les auteurs de cet amendement, la création du CSE se traduirait par un recul des prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail, pour la seule raison que ne sont pas reprises mot pour mot les dispositions antérieures relatives au CHSCT. Or cette réforme prend également la forme d'un grand exercice de réécriture de plusieurs centaines d'articles du code du travail. Certains aspects ont été mis en facteur commun au sein d'un article socle rassemblant les principales attributions du CSE, qui sont détaillées ensuite. C'est le cas notamment de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, qui est désormais mentionnée à l'article L. 2312-5, l'article L. 2312-6 disposant que ses attributions sont étendues en la matière aux salariés mis à disposition. Je tiens par ailleurs à vous faire remarquer que, lorsque les membres du CSE constatent que l'employeur ne se conforme pas à ses obligations légales en matière de santé et de sécurité, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Ainsi, en cas de danger grave et imminent, ils peuvent, par le biais

les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle », selon l'article L. 2312-5 du même code. Il s'agit cette fois

vote. Madame la ministre, je crois que nous avons, là encore, une divergence de fond.

les problèmes de santé et de sécurité

repris dans l'ordonnance n° 2017-1386. Nous l'avons déjà évoqué lors de l'examen de l'article 2, la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est primordiale. Or nous trouvons qu'elle est insuffisamment traitée dans

Nous proposons ici de préciser concrètement les informations que devrait, selon nous, comporter la base de données économiques et sociales. En effet, en l'état actuel du texte, cela reste très flou, puisqu'il n'est fait état que des écarts de rémunération, ce qui est certes important, mais loin d'être le seul sujet en la matière.

en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. l'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, les données relatives à l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, ainsi qu'à la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration. Je ne suis pas persuadée, au moment où je vous parle, que ce

L'ordonnance n° 2017-1386 se borne en effet à proposer la présence « d'indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les écarts de rémunération. » Compte tenu de l'importance de ce problème et de l'engagement du Gouvernement dans une politique de renforcement des obligations des entreprises en matière d'égalité professionnelle, la mention précise des indicateurs à renseigner

commission ? Comme on l'a beaucoup répété depuis maintenant plus de six mois et l'ouverture des débats sur la loi d'habilitation, l'un des objectifs de cette réforme est d'élargir le champ de la négociation d'entreprise à des domaines qui lui étaient jusqu'à présent fermés, afin de laisser aux partenaires sociaux, en son sein, la possibilité d'adapter par accord, c'est-à-dire s'ils parviennent à un compromis, le cadre légal aux particularités de l'entreprise. À défaut d'accord, des dispositions supplétives, strictement identiques au droit antérieur, s'appliquent. L'un des domaines nouvellement ouverts à la négociation est celui du contenu de la base de données économiques et sociales, la BDES, qui doit être alimentée par l'employeur et fournir aux représentants du personnel les informations dont ils ont besoin pour rendre leurs avis lorsqu'ils sont consultés.

En l'absence d'accord sur la BDES, ces dispositions trouveront bien à s'appliquer. En revanche, si les syndicats majoritaires dans l'entreprise estiment que certaines des informations mentionnées ici ne sont pas pertinentes dans leur cas particulier, mais que d'autres indicateurs le seraient davantage, il faut leur faire confiance. Par ailleurs, cet amendement tend un rapport de situation comparée sur support papier faisant référence au comité d'entreprise et aux délégués du personnel sans tenir compte de la création du CSE. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

le plus important est que les partenaires sociaux se saisissent du sujet. Il est vrai qu'il n'y a pas d'accord ou de plan d'action partout, alors que c'est obligatoire. De plus, la qualité du contenu et le degré d'engagement des accords sont assez inégaux.

M. Daniel Chasseing. Dans le cadre de la base de données économiques et sociales, ou BDES, les entreprises sont parfois amenées à fournir des informations qui ont un caractère confidentiel. Le code du travail garantit le respect du devoir de discrétion des représentants du personnel. Néanmoins, la protection des données n'est pas assurée au niveau des fournisseurs de logiciels de bases de données « clef en main » qui peuvent être amenés

mais partent du postulat qu'un hébergeur situé à l'étranger serait par nature moins fiable qu'un hébergeur français ou européen. Or ceux-ci peuvent tout autant être les victimes de piratages ou même d'employés indiscrets ou malveillants.

monsieur le président.

est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à revenir sur l'une des principales modifications

dans le cadre de la loi Rebsamen, ces consultations concernent trois grands domaines : orientations stratégiques de l'entreprise ; situation économique et financière ; politique sociale, conditions de travail et emploi. Elles doivent en principe avoir lieu tous les ans. L'ordonnance a ouvert aux partenaires sociaux dans l'entreprise la possibilité de modifier cette périodicité, dans la limite de trois ans. Je ne partage pas les réticences des auteurs de cet amendement, qui estiment que cet élargissement du champ du dialogue social lui serait néfaste au contraire, il responsabilise les organisations syndicales et l'employeur. Par exemple, est-il nécessaire d'examiner tous les ans dans toutes les entreprises leurs orientations stratégiques ? Les entreprises dotées d'un plan pluriannuel de développement et de production ne trouveraient-elles pas intérêt à y procéder tous les deux ou trois ans, pour consacrer dans ce cas, peut-être, plus de temps aux consultations sur la politique sociale et aux enjeux relatifs aux conditions de travail ? Il ne faut pas restreindre le champ du dialogue social ou considérer que ses acteurs en entreprise ne pèsent pas les conséquences des accords qu'ils La commission a donc émis un avis défavorable

le recadrer : c'est une négociation annuelle sur la base d'une réflexion pluriannuelle, ce qui oblige à remettre le sujet sur la table

la législation et de remettre de l'ordre et de la transparence dans les transactions financières internationales. Il convient également d'exiger la transparence des multinationales et la disparition des sociétés-écrans et des prête-noms. Pour remplir ces objectifs, il faut renforcer les moyens humains et matériels des administrations fiscales, mais aussi renforcer les pouvoirs de contrôle des salariés dans les domaines économiques et financiers et, plus particulièrement, en matière fiscale et sociale. proposons donc de permettre au comité d'entreprise d'être informé et consulté sur la politique de prix de transferts retenue par l'entreprise et sur les cessions d'actifs réalisées au sein d'un même groupe.

Face aux politiques fiscales pratiquées par certains de ces grands groupes, il y a lieu d'instaurer un droit leur faisant contrepoids. tend donc à octroyer aux représentants des salariés un droit de regard sur la politique fiscale de leur entreprise en consolidant la procédure d'information et de consultation sur ce thème et en offrant la possibilité de recourir, dans certains cas, à un expert

puisque la base de données économiques et sociales doit déjà contenir des informations relatives aux « transferts commerciaux et financiers » entre les entités d'un groupe. S'agissant de la politique fiscale de l'entreprise, elle doit relever exclusivement de l'employeur : il n'appartient pas aux représentants des salariés

en matière économique et saisir de cette question le conseil d'administration ou de surveillance. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement

Ensuite, dans bien des cas, on découvre, quand la filiale française est déjà en train de fermer ou est en faillite, que c'est par un mécanisme de prix de transfert que l'on l'a vidée de sa substance pour la mettre artificiellement en déficit.

L'entreprise est commune aux salariés qui travaillent et aux dirigeants qui prennent les décisions. Malheureusement, la séparation des tâches entre la prise de décision et son application ne permet pas aux salariés de s'impliquer réellement.

en reconnaissant aux représentants du personnel un droit de vélo suspensif sur les décisions de l'employeur relatives à des projets de restructuration de l'entreprise ou de compressions d'effectifs : délocalisations, licenciements collectifs, transferts de production de moyens de production d'un établissement à un autre, de la même entreprise ou du même groupe. Il nous semble vital que les salariés, par leurs représentants, puissent non seulement donner leur avis, mais aussi décider lorsque les sujets intéressent directement la gestion de l'entreprise : organisation du travail, formation professionnelle, gestion économique et financière. L'entreprise étant un bien collectif, il paraît nécessaire d'en moderniser la gouvernance. Si votre projet de loi vise réellement à mieux partager les pouvoirs dans les entreprises, madame la ministre, il n'y a aucune raison d'exclure du nouveau cadre de relations entre salariés et employeurs les choix économiques qui ont trait à la vie de l'entreprise. Quel est l'avis de la commission ? Selon les auteurs de cet amendement, l'employeur devrait suspendre ses projets de restructuration sur injonction du CSE, s'il n'a pas suffisamment pris en compte les remarques de ce dernier. L'objet de cette réforme du droit du travail n'est pas d'instaurer la cogestion des entreprises. Néanmoins, elle ouvre la possibilité, par accord d'entreprise, de transformer le CSE en conseil d'entreprise doté d'un droit de veto dans les domaines que cet accord aura définis.

au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Dans la mesure où ces sommes sont issues de la plus-value réalisée par les salariés, il est normal de les mettre à contribution en faveur des activités sociales et culturelles de l'entreprise. Quel l'avis de la commission ? l'ordonnance rompait avec le droit antérieur en élargissant cette assiette, qui correspondait à la masse salariale, aux sommes versées dans l'année au titre de l'intéressement et de la participation. Une brève brève réflexion sur les conséquences néfastes de cette mesure ne peut que nous conduire à la supprimer, ce que nous avons fait en commission. En effet, elle a un caractère désincitatif très fort pour les entreprises en matière de développement de l'intéressement et de la participation. À l'heure où le Gouvernement a fait part de son intention de développer l'épargne salariale, les entreprises déjà engagées dans ces pratiques seraient sanctionnées par une augmentation potentiellement très importante de leur contribution financière aux activités sociales et culturelles, tandis que celles qui y étaient jusqu'à présent réticentes verraient leurs craintes renforcées. Il n'est donc pas souhaitable, sur ce point, de revenir au texte d'origine. Je ne doute pas que Mme la ministre sera d'ailleurs de mon avis sur cette question. Par ailleurs, cet amendement ne vise pas le bon alinéa,

de l'entreprise à établissements multiples sont au moins égaux à 50 salariés. En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 2313-1 du code du travail laisse entendre que, dès lors qu'une entreprise comporte au moins deux établissements distincts,

comprenant des établissements distincts. Les articles L. 2316-1 à L. 2316-3 fixent les attributions d'un CSE d'une entreprise d'au moins 50 salariés. Par conséquent, un CSE central dans une entreprise de moins de 50 salariés comportant des établissements ne disposerait pas d'attributions. CQFD ! La vigilance du Sénat est précieuse, et je vous en remercie.

que le Sénat a exprimée dès 2015 lors de l'examen de la loi Rebsamen : les suppléants ont vocation à remplacer les titulaires en cas d'absence, et non à être présents à leurs côtés en permanence, puisqu'ils n'ont aucune attribution propre.